d’observation ?… Le procès verbal est adopté sous les réserves d’usage. L’ordre du jour appelle le débat à la suite du dépôt du rapport public annuel de la Cour des comptes.

Il s’agit d’un rendez vous important, car il nous apporte un éclairage précieux pour l’exercice de notre mission constitutionnelle de contrôle de l’action du Gouvernement. Vos conclusions et les orientations qui les accompagnent nourrissent également nos débats législatifs. Je vous remercie donc de votre présence, mais aussi

Comme chaque année, je donnerai la parole aux présidents de la commission des finances et de la commission des affaires sociales, puis à un représentant de chaque groupe politique, afin que le Sénat puisse s’exprimer, dans toute sa diversité, sur les observations et recommandations formulées dans ce rapport public annuel.

En tout état de cause, il reste, vous le soulignez, des défis à relever. Au premier rang de ces défis figurent les disparités territoriales – nous venons d’échanger à ce sujet –, qui affectent notamment

une chance et une source d’immenses défis. Les politiques conduites en ce domaine ne sont pas seulement une réponse à des besoins immédiats ; elles sont aussi un investissement stratégique visant à bâtir une société plus résiliente, plus prospère et plus équitable. La jeunesse

Les politiques publiques en faveur des jeunes sont un enjeu massif en matière de dépenses publiques. La Cour a calculé le montant des dépenses de l’État spécifiquement destinées aux jeunes âgés de 15 à 25 ans : nous les avons estimées à 53,4 milliards d’euros, soit 12 % du budget de l’État et 2 % du PIB

à l’enseignement supérieur. Je dirai quelques mots de l’orientation au collège et au lycée. Malgré l’importance de l’enjeu et malgré son coût, qui est de quelque 400 millions d’euros, cette politique ne permet pas pas de dépasser les déterminismes, les stéréotypes et les inégalités entre filières. La Cour préconise notamment de rendre obligatoires des modules relatifs à l’orientation dans la formation initiale des enseignants, qui sont désormais chargés de cette mission avec les régions, et d’adapter leurs emplois du temps pour qu’ils assument pleinement cette compétence. J’aimerais également insister que nous avons consacrée à l’accès des jeunes ruraux à l’offre d’enseignement supérieur. J’ai déjà dit les chiffres : nous constatons que les jeunes ruraux accèdent beaucoup moins fréquemment

en veillant au partage d’expériences entre territoires, grâce à la désignation d’un chef de file à l’échelon national. L’emploi comme le logement impliquent parfois une mobilité géographique importante, en particulier pour les jeunes situés dans les zones rurales ou périurbaines. C’est pourquoi j’aimerais également vous livrer certains de nos constats sur la mobilité des jeunes en transports collectifs. 38 % des jeunes ruraux ont déjà renoncé à un entretien d’embauche en raison de difficultés de déplacement. Les autorités organisatrices de la mobilité ont pour stratégie d’octroyer aux jeunes des réductions tarifaires, sans cibler les plus défavorisés et au prix de pertes de recettes. Or c’est non pas le prix, mais plutôt le manque d’offre, notamment dans les zones périurbaines et rurales, qui entrave la mobilité des jeunes. Nous préconisons donc d’améliorer la connaissance de ce dont ils ont besoin pour se rendre au travail, de mieux tenir compte des ressources dans l’octroi d’avantages tarifaires et de mieux coordonner l’offre entre collectivités. J’en arrive à la troisième partie du rapport, où sont examinées les politiques de prévention à destination de la jeunesse, qu’il s’agisse d’encourager les pratiques sportives, de prévenir les addictions ou de lutter contre les mauvaises habitudes alimentaires.

des pratiques sportives entre 15 et 25 ans. En outre, les politiques publiques s’adressent davantage aux jeunes déjà sportifs qu’aux profils les plus éloignés d’une pratique, comme les femmes, les jeunes en situation de handicap ou ceux qui sont en difficulté socio économique. Ces profils devraient être les cibles d’une stratégie définie et mise en œuvre par l’État en lien avec les collectivités et les acteurs privés du sport.

ils ont été brouillés par la pluralité des messages. Le ministre des armées a récemment annoncé une nouvelle réforme de la JDC visant à la remilitariser. Il faudrait en profiter pour rationaliser les objectifs, le contenu et la base juridique du dispositif, au moment où il est essentiel de renforcer le lien entre les jeunes, la Nation et l’armée.

12 % de la population française, mais 26 % des mis en cause, 34 % des poursuivis et 35 % des condamnés en 2023.

c’est que le problème tient non pas à la quantité de la dépense – la jeunesse française n’est pas abandonnée par l’État et les acteurs publics –, mais à sa qualité

mieux différencier les soutiens et les mesures en fonction des publics ciblés. Tous les jeunes ne disposent pas des mêmes chances. Les politiques publiques doivent réduire les inégalités en passant d’un pilotage par l’offre

La jeunesse – nous l’avons vécue – est un moment passionnant, mais intrinsèquement délicat et parfois difficile. La plupart des politiques en faveur de la jeunesse ont intégré cette dimension.

Monsieur le président, monsieur le Premier président,

que nous leur avions demandée sur la gestion de l’eau potable et de l’assainissement en outre mer. Plus largement, les rapporteurs spéciaux de la commission suivent avec attention les travaux de la Cour des comptes, chacun dans leur domaine de compétences.

Je ne reviendrai pas sur les conclusions de notre mission d’information sur la dégradation des finances publiques depuis 2023, sauf peut être pour rappeler que celles ci ont été adoptées à l’unanimité, ce qui ne sera peut être pas le cas sur Je me contenterai d’indiquer l’objectif du Gouvernement pour la préparation du budget pour 2026 : réduire le déficit public de 5,4 % à 4,6 % du PIB, tout en augmentant les dépenses d’investissement dans l’industrie de défense et en préservant notre modèle social. Cette équation ferait sans doute peur à plus d’un mathématicien ; la porte parole du Gouvernement a d’ailleurs elle même parlé hier de « cauchemar » ! Difficile d’employer un terme plus fort… Seul point positif dans ce tableau, les comptes nationaux des administrations publiques présentés ce matin par l’Insee font apparaître, pour 2024, un déficit inférieur à à la prévision, de 5,8 % du PIB, ce qui signifie que, malgré une croissance probablement plus faible que ce qui était espéré pour 2025, la marche des 5,4 % de déficit reste atteignable. J’en reviens au cœur de ce rapport public annuel.

Pierre Bourdieu disait, dans une formule restée célèbre, que « la “jeunesse” n’est qu’un mot », pour souligner que, derrière l’apparente uniformité d’une génération, se cachent en réalité des situations radicalement différentes et, pour le dire sans détour, de profondes inégalités. la Cour n’ignore pas cette difficulté et la prend au contraire à bras le corps, en montrant avec précision et clarté que tous les jeunes n’ont pas les mêmes chances selon le lieu où ils vivent,

Le défi est considérable. Un jeune sur dix vit sous le seuil de pauvreté, contre 7,7 % des 26 65 ans, et la santé mentale des jeunes s’est fortement dégradée au cours des dernières années. Nous avons tous une responsabilité à l’égard de la jeunesse de notre pays. Je me réjouis donc que la Cour des comptes ait décidé cette année de faire un bilan des politiques menées dans ce domaine. L’accès aux moyens de transport collectif joue un rôle

Or la Cour remarque que le principal frein à la mobilité des jeunes tient moins au tarif qu’à l’offre de transport disponible. Sur l’initiative de la commission des finances, l’une des principales recommandations

affectés par an aux AOM. Ce montant, il faut le dire, reste modeste, mais il s’ajoute à l’enveloppe existante et traduit une orientation qui doit être poursuivie.

tandis que 48 % des jeunes en situation de non emploi résident toujours chez leurs parents cinq ans après la fin de leurs études ». L’accès au logement des jeunes à la recherche de leur premier emploi demeure un angle mort

alors que les jeunes non étudiants sont majoritaires au delà de 21 ans. Il s’agit bien entendu non pas d’opposer les catégories entre elles, mais de faire en sorte que la politique du logement réponde plus efficacement aux besoins.

même si ce taux reste deux fois supérieur à celui de la population générale. L’effort financier de l’État en faveur de l’emploi des jeunes est indéniable : les dépenses publiques ciblées sont passées de 3,4 milliards d’euros en 2017 à 7,2 milliards d’euros en 2023, principalement sous l’effet de la montée en puissance des aides à l’apprentissage. Toutefois, la Cour relève que le lien de causalité entre les deux phénomènes n’est pas entièrement établi et que le principal déterminant de l’accès des jeunes à l’emploi demeure la conjoncture économique. Les magistrats financiers préconisent donc une stratégie qui privilégie les politiques contracycliques et notent que le maintien de la dépense à un à un niveau très élevé depuis 2022 ne répond pas à cette logique. Lors de l’élaboration de la loi de finances pour 2025, la commission des finances avait également plaidé pour un recentrage de ces aides sur les jeunes les plus éloignés de l’emploi. à présent mon propos sur deux politiques plus sectorielles, mais qui ont une réelle importance : la prise en charge des jeunes majeurs issus de l’aide sociale à l’enfance et l’orientation des jeunes. La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite loi Taquet, a créé un droit opposable à l’accompagnement des jeunes majeurs issus de l’aide sociale à l’enfance.

La mise en œuvre de cette loi est toutefois encore très partielle et varie fortement d’un territoire à l’autre. L’effort financier des départements, lui aussi, reste inégal. L’une des raisons est la faiblesse de la compensation financière allouée par l’État au regard du coût de la politique. Une enveloppe de seulement 50 millions d’euros par an y est consacrée, alors même que le montant des dépenses est estimé à 1,2 milliard

se disent insatisfaits des informations et des conseils qu’ils reçoivent dans leur établissement. L’orientation demeure en outre genrée et inégalitaire : les filles ne représentent que 13,7 % des effectifs de terminale professionnelle avec des spécialités de production. Seuls 62,1 % des élèves des zones rurales éloignées choisissent une seconde générale et technologique, contre 76,4 % des élèves des zones urbaines denses.

pour ce tour d’horizon très complet et pour les recommandations assorties. Il nous sera précieux pour nos analyses, notamment lors de la préparation des prochains textes financiers, afin de définir la meilleure allocation possible des moyens

l’emploi des jeunes et les difficultés spécifiques que ceux ci rencontrent en matière d’insertion professionnelle. Les moyens mis en œuvre en faveur de cette population ont été doublés depuis 2017, pour atteindre 7,3 milliards d’euros en 2023. Pour autant, les statistiques de l’accès à l’emploi sont connues et, en dépit de réelles améliorations depuis 2018, le taux de chômage chez les jeunes demeure de 17,2 % en 2023, soit un niveau 2,4 fois plus élevé que celui de l’ensemble des actifs. L’enquête menée par la Cour permet d’objectiver un constat : augmenter la dépense publique n’est pas un gage de meilleurs résultats. Plus précisément, rien ne semble assurer que l’amélioration relative de l’emploi des jeunes soit la conséquence de l’effort financier consenti par les pouvoirs publics. La conjoncture économique reste le premier déterminant de l’accès des jeunes à l’emploi. Aussi paraît il urgent de revoir la stratégie en faveur de l’emploi des jeunes. À cet égard, le dispositif « 1 jeune, 1 solution », pertinent pour répondre à la crise sanitaire, ne peut être indéfiniment prolongé.

Vos recommandations rejoignent les nôtres sur ce point. Enfin, vous vous intéressez aux évolutions du contrat d’engagement jeune (CEJ) résultant de la loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023. Le rapprochement des missions locales et de France Travail a abouti à un équilibre fragile, entre complémentarité et concurrence dans l’accompagnement des jeunes. Plus généralement, la piste évoquée d’une réduction du nombre de contrats pour les recentrer sur les jeunes les plus éloignés de l’emploi nous semble prometteuse et propre à concilier efficacité de la dépense publique et accompagnement renforcé des publics les plus en difficulté. L’enquête de la Cour traite également d’un autre sujet de grande importance : l’aide sociale à l’enfance et, plus précisément, la prise en charge des jeunes majeurs qui en sont issus. La loi du 7 février 2022 a renforcé les missions du département en matière d’accompagnement des jeunes majeurs pour mettre fin aux situations de sortie sèche du système de protection de l’enfance, Elle rend obligatoire de proposer une solution aux jeunes sortant de l’ASE jusqu’à leurs 21 ans lorsqu’ils ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.

Malgré cette légère baisse, le coût, comme vous l’indiquez, a augmenté pour s’établir à 1,2 milliard d’euros en raison d’une hausse des mesures d’accueil, plus coûteuses. Pourtant, la prise en charge des jeunes majeurs à leur sortie de l’ASE reste le parent pauvre des politiques de protection de l’enfance. Ainsi, l’État a débloqué en 2022 une enveloppe de seulement 50 millions d’euros à ce titre, répartie simplement au prorata des jeunes pris en charge et sans condition de respect de certaines exigences par les départements. donc le delta qui sépare l’engagement de l’État et les obligations des départements… Par ailleurs, comme vous le relevez, malgré quelques améliorations, les dispositifs prévus par la loi de 2022 sont encore loin d’être pleinement appliqués les commissions départementales d’accès à l’autonomie des jeunes majeurs sont absentes de nombreux départements et l’entretien bilan six mois après la fin du contrat jeune majeur n’est que trop rarement réalisé, faute, je le répète, de moyens d’accompagnement des départements. Je relève tout particulièrement votre inquiétude, déjà identifiée par notre commission, concernant les disparités territoriales dans la prise en charge par l’ASE. Ainsi, la Cour relève que le taux de prise en charge des jeunes majeurs varie de 38 % seulement en Seine et Marne à 83 % en Gironde Nous ne pouvons que regretter l’absence de pilotage de l’ensemble de la dépense. Je note enfin une faiblesse majeure dans le dispositif de suivi des jeunes majeurs en situation de handicap.

La Cour des comptes, par ailleurs, a consacré un chapitre aux addictions des jeunes aux drogues illicites et à l’alcool, addictions dont les conséquences sanitaires, sociales et économiques sont lourdes. La situation est préoccupante à plus d’un titre. Malgré une baisse sensible des niveaux de consommation d’alcool et de drogues illicites chez les mineurs, les données restent élevées chez les jeunes majeurs. Vous le montrez bien : au sein de l’Union européenne, la France se démarque, aujourd’hui encore, par des indicateurs très défavorables, qu’il s’agisse de la fréquence de la consommation quotidienne d’alcool ou des niveaux d’usage de drogues illicites, notamment de cannabis et de cocaïne. Face à cette situation, qui reflète notamment un déficit de prévention auprès des jeunes, la réponse sanitaire et médico sociale actuelle est à la fois insuffisante et inadaptée. En matière de dépistage, d’abord, des carences majeures sont à déplorer en raison d’un déficit de formation des médecins généralistes. En ville, deux tiers d’entre eux déclarent ne pas connaître les démarches de repérage précoce. pour la prise en charge, les jeunes se tournent peu vers les centres d’accompagnement, alors que ces structures spécialisées devraient constituer un relais de la prévention et de l’accompagnement. Quant à l’offre hospitalière, elle est à la fois très en deçà des besoins et peu ciblée sur les adolescents et les jeunes adultes. Les consultations jeunes consommateurs représentent aujourd’hui l’unique dispositif spécifiquement consacré à l’accueil des jeunes. Au nombre de 260, ces structures souffrent néanmoins d’un sous dimensionnement notoire. La commission des affaires sociales souscrit à la recommandation de bâtir une politique de prévention plus ambitieuse et souligne la nécessité de la prolonger par un système de prise en charge mieux coordonné.

Nous partageons les préoccupations de la Cour des comptes et sa recommandation de clarifier les missions qui demeureront affectées à cette journée. Nous avons d’ailleurs soutenu cette logique lors de l’examen du projet de loi de finances. Comme la Cour le souligne, il conviendra d’aller au bout de cette démarche et de déterminer ce que nous souhaitons faire de cette journée. Quelques heures ne peuvent suffire à insuffler l’esprit de défense, à dispenser un enseignement civique, à détecter l’illettrisme et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes… Si ce débat était mené à terme, il faudrait en tirer les conséquences dans un texte encadrant la JDC. Le rapport confirme, par ailleurs, que la mise en place du service national universel (SNU) a perturbé l’organisation de cette journée.

Là encore, nous pensons qu’il faut engager une réflexion globale sur les dispositifs en faveur de la jeunesse qui promeuvent le lien entre l’armée et la Nation ou qui prodiguent des enseignements à la citoyenneté.

Cette année, monsieur le Premier président, vous avez sondé directement les politiques publiques en faveur des jeunes. Vous avez analysé de nombreux dispositifs destinés à la jeunesse pour étudier leur efficacité,

Pour autant, lorsqu’on étudie le détail de ce résultat et la répartition des diplômés sur le territoire, les chiffres sont beaucoup moins bons. Près d’un tiers de la population française – 32 % – est diplômée de l’enseignement supérieur, quand ce taux s’établit

des centres de formation d’apprentis gérés par les chambres consulaires. Par ailleurs, le développement de l’offre d’enseignement supérieur dans ces territoires est rendu difficile par le déclin démographique qui y a cours. Comme pour beaucoup d’autres politiques publiques, la solution doit venir d’une redynamisation des territoires ruraux, qui ont longtemps été abandonnés par l’État. Il faut redonner à nos jeunes les mêmes espoirs et les mêmes perspectives que ceux dont jouissent leurs camarades des grandes villes. Les solutions sont nombreuses : réindustrialiser pour créer des emplois durables, construire des logements adaptés aux besoins de la population, développer une véritable offre de transport en commun permettant d’aller étudier et travailler, et garantir

l’accompagnement de nos jeunes. J’en retiens trois, qui me paraissent devoir être mises en œuvre rapidement. Tout d’abord, vous préconisez d’adapter l’emploi du temps des professeurs principaux pour leur permettre d’assurer leur mission d’orientation des jeunes. Ensuite, vous appelez à rendre plus accessibles et lisibles les dispositifs

un maquis d’aides et de dispositifs. Ce phénomène, encore amplifié dans les territoires ruraux, est regrettable. Un point de ce rapport attire particulièrement mon attention

Les politiques publiques en leur faveur ne sont pas seulement une réponse à des besoins immédiats. Elles constituent aussi un investissement stratégique pour bâtir une société plus équitable, résiliente et prospère. En accompagnant cette période charnière de la vie, ces politiques permettent à chaque jeune de réaliser son potentiel tout en renforçant la cohésion sociale et le progrès collectif. » Monsieur le Premier président, le groupe RDPI vous remercie d’avoir choisi Dans un contexte mondial marqué par des transformations économiques et géopolitiques rapides ainsi que par des enjeux environnementaux croissants, il est essentiel de doter notre jeunesse des outils nécessaires pour relever ces défis.

D’autres acteurs interviennent également, comme les collectivités locales ou les organismes de sécurité sociale. Il en résulte une prolifération de dispositifs qui finit par rendre illisibles et complexes certaines de ces politiques, ce qui nuit à leur efficacité. Ainsi, de nombreux jeunes ne font pas appel aux programmes auxquels ils ont droit et ce sont malheureusement souvent ceux qui en ont le plus besoin. En matière d’éducation, nous pourrions, au premier abord, nous féliciter du grand nombre de diplômés de l’enseignement supérieur : plus de la moitié de la génération sortie d’études en 2021, soit davantage que la moyenne européenne. situation cache d’importantes disparités régionales : les grandes métropoles font beaucoup mieux que les territoires ruraux ou ultramarins. Dans le même temps, nous sommes également au dessus de la moyenne européenne nombre de jeunes en difficulté ou à faible compétence. Notre système éducatif reste très inégalitaire, avec des propositions d’orientation scolaire souvent influencées par le genre et l’origine sociale ou territoriale, ce qui laisse de côté une partie des jeunes, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. La transition vers la vie active peut également être difficile. Trop de jeunes peinent à s’insérer durablement sur le marché du travail et les freins à la mobilité accentuent ces difficultés. Pour autant, globalement, le chômage des jeunes connaît une baisse continue, ce qui traduit une réussite des politiques dans ce domaine. La généralisation de l’alternance est un progrès. Il nous faut toutefois, au regard de son coût, mieux la cibler et aller plus loin en multipliant les passerelles vers l’emploi durable et en adaptant nos dispositifs aux spécificités locales. Justement, les outre mer présentent nombre de ces spécificités et concentrent beaucoup des problèmes recensés.

si nationalement ce taux baisse, il stagne depuis des années en outre mer, et il augmente même en Guyane. Par ailleurs, l’illettrisme y est massif : de 30 % à 50 % des jeunes sont concernés, et la moitié d’une classe d’âge quitte le système scolaire sans diplôme autre que le brevet des collèges. Quel avenir pour des territoires où la jeunesse est si mal formée ? Autre réalité spécifique aux outre mer : beaucoup de jeunes quittent leur territoire d’origine pour se former, mais, faute de perspective professionnelle, c’est un départ sans retour. Ce mouvement dramatique pèse sur l’équilibre démographique, notamment aux Antilles, où la natalité ne compense pas cette perte. Il appauvrit globalement le territoire, avec une fuite des compétences souvent irréversible. mes chers collègues, à prendre connaissance du rapport sur la jeunesse ultramarine de Rodolphe Alexandre, ancien président de la collectivité territoriale de Guyane, remis voilà tout juste un an à Marie Guévenoux, alors ministre déléguée chargée des outre mer. Ses conclusions et recommandations sont proches de celles du rapport annuel de la Cour des comptes, notamment sur l’éparpillement et la superposition des aides et le non recours. Enfin, je dirai un mot sur les problématiques liées à la santé. d’addictions, de santé mentale, d’obésité et de précarité alimentaire, qui touchent une proportion inquiétante de jeunes, peuvent avoir des répercussions tout au long de leur vie. Une prise en charge précoce, avec des parcours de soins adaptés, est donc primordiale. Mais plus encore, nous devons avoir la volonté de mettre en place une politique de prévention ambitieuse. C’est particulièrement frappant pour ce qui concerne les addictions. La consommation de drogues illicites et d’alcool est très élevée en France, au dessus de la moyenne européenne. C’est un constat d’échec de notre politique. Le rapport évoque les pays du nord de l’Europe, comme le Danemark et l’Islande, qui ont montré qu’il était possible de faire baisser les consommations de manière importante par la prévention. Nous devons nous en inspirer et faire évoluer notre approche, aujourd’hui presque exclusivement répressive. Notre incapacité à faire baisser la consommation de drogues a une incidence directe sur la réussite de nos politiques publiques. La criminalité liée aux trafics pour alimenter les consommateurs attire une frange attire une frange de notre jeunesse, la détourne de l’éducation et la fait plonger dans la délinquance. Les territoires d’outre mer qui se trouvent sur les nouvelles routes de ce trafic mondial paient déjà un lourd tribut. Pour conclure, je remercie la Cour des comptes pour ce travail d’importance qui vient éclairer les failles de nos politiques à destination de la jeunesse. Des progrès restent à accomplir pour surmonter la persistance des inégalités et du déterminisme social.

la Cour des comptes consacre son rapport public annuel 2025 aux politiques publiques en faveur de la jeunesse. C’est un excellent choix, car le débat public se concentre trop souvent sur la question des retraites plutôt que sur celle de la réussite de notre jeunesse, qui incarne pourtant l’avenir de notre pays. La période actuelle ayant des relents de guerre de plus en plus palpables, la paix est un horizon à reconquérir et l’hypothèse du retour de la conscription revient dans les débats. Dans ce contexte, il est réjouissant de que 50 % des jeunes de 18 à 30 ans seraient prêts à s’engager en cas de conflit – beaucoup plus qu’aux Pays Bas ou en Allemagne – et que les candidats à la réserve citoyenne se bousculent.

Un chapitre du rapport traite de l’apprentissage de la citoyenneté. C’est pour moi le cœur du sujet. Ce n’est pas à 15 ou 18 ans que l’on apprend la République et le respect des règles du vivre ensemble. Tout se joue dès la prime enfance, dès l’école maternelle et primaire. Une métaphore paysanne s’impose. Quand un vigneron met un tuteur à un pied de vigne, il faut le planter très tôt. Si l’on attend que le cep soit adulte, c’est trop tard. Il en va de même pour l’efficacité des politiques publiques pour la jeunesse. L’école ne peut pas tout et, malgré ses efforts, son action ne porte que sur quatre jours par semaine et trente six semaines par an. Comment renouer avec les 10 % de jeunes exclus de l’emploi, avec ceux qui tombent dans la délinquance,

d’ailleurs porté, monsieur le Premier président, un regard sévère sur ce dispositif. Victor Hugo invitait la République à favoriser chez les jeunes « un authentique savoir être citoyen » et à recréer les conditions qui permettent d’élever « l’homme à la dignité de citoyen ». Je propose d’innover en instaurant une nouvelle forme de tutorat pour tous les enfants dès l’âge de 3 ans, dès l’école maternelle. Reste à inventer la forme de ce dispositif qui devrait, selon moi, réunir l’école et la mairie, ces deux socles de notre République. Cette mesure permettrait de renforcer l’adhésion précoce à la citoyenneté, de réduire les inégalités sociales, de prévenir l’échec scolaire et la petite délinquance, mais sans tomber dans une vision « bisounouresque

En conclusion, je me réjouis que ce débat sans posture, sans dogmatisme, démontre une fois de plus la qualité du travail de notre assemblée. Je vous remercie, monsieur le président, d’avoir organisé ce débat. La parole

merci.

Pascal Savoldelli. Monsieur le président, monsieur le Premier président de la Cour des comptes, mes chers collègues, la jeunesse est le miroir de notre société. Elle est plurielle, fragmentée, traversée de tensions et de luttes. Elle partage une même volonté : l’accès à l’éducation, à l’emploi, au logement, à l’autonomie. Le rapport de la Cour des comptes nous rappelle la gravité de la situation de cette classe d’âge, notamment en termes de précarité et de souffrance psychologique. Qui peut ignorer ces files d’étudiants devant les Restos du Cœur ou l’augmentation inquiétante des troubles mentaux chez les 18 24

Car ce mal être est autant social que politique : il trouve sa source dans les échecs ou les renoncements des différentes majorités gouvernementales. Le néolibéralisme a fait de la jeunesse le cheval de Troie de la flexisécurité, le laboratoire d’une société déshumanisée où les contrats précaires, les stages interminables et l’ubérisation du travail sont devenus, pour trop de jeunes, la norme. L’accès à un travail digne, stable et rémunéré semble de plus en plus inatteignable. Ce système, qui recourt au discours de l’« employabilité » pour justifier l’exploitation et la précarisation, n’a que trop duré. On teste, on dérégule, on met en concurrence… Après Parcoursup, cette brutalité sociale se retrouve aussi sur le marché du travail

Territorialement, la fracture s’aggrave : 14 % de chômage en plus pour les jeunes des quartiers populaires, 22 % pour les jeunes ruraux. Aujourd’hui, un nombre croissant de jeunes s’engagent

Cette dynamique ne se résume pas à une simple réaction face à la précarité. Elle incarne une véritable volonté de changer la société. En témoigne le rejet croissant du système capitaliste, responsable de la crise climatique et des inégalités croissantes. (Ifop), en 2023, 60 % des jeunes considéraient que le capitalisme était le principal responsable de cette crise et 64 % d’entre eux aspiraient à un monde plus solidaire et équitable. Cette aspiration ne se limite pas à un rejet du système en place. Il s’agit aussi de proposer une alternative : une éducation réellement démocratique, non soumise aux impératifs du marché. Le néolibéralisme a transformé l’éducation en une simple préparation à l’intégration dans le marché du travail, mais il nous revient de repenser l’éducation comme un outil d’émancipation. Ayons l’ambition de transformer l’école en une « institution du commun », contrôlée démocratiquement par les usagers, les professionnels et la population. Nous devons abolir la concurrence entre établissements, éradiquer la ségrégation ethnique et sociale, repenser l’inclusion. Il s’agit non pas seulement de défendre une école d’État face à une école de marché, mais de repenser cette école afin qu’elle soit véritablement un vecteur d’égalité, de justice sociale et de solidarité. Repenser l’école, c’est aussi interroger la jeunesse sur son rapport au travail. Quel monde du travail préparons nous ? Produire quoi ? Pour qui ? Dans quelles conditions ? Il est temps d’affirmer une autre vision, celle d’un travail libéré du chantage à l’emploi, reconnu pour sa valeur sociale et non pour sa rentabilité immédiate. Grâce à vos travaux, monsieur

Monsieur le président, monsieur le Premier président, mes chers collègues, cette année, le rapport annuel de la Cour des comptes nous pose, au travers de ses plus de 600 pages, une question simple chaque jeune Français, quels que soient son lieu de naissance, son genre ou son origine sociale, a t il les mêmes opportunités qu’un autre pour construire son avenir ? On parle de 2 % du PIB et de 12 % du budget de l’État dédiés à la jeunesse

avec pour conséquence de limiter les ambitions des jeunes. Plus grave, et ce point doit interpeller la chambre des territoires, les inégalités territoriales demeurent très importantes dans l’accès à une solution de formation, malgré la loi de 2018. une véritable rupture d’égalité pour la jeunesse des territoires ruraux. Le taux de diplômés de l’enseignement supérieur varie selon les régions et diminue à mesure que l’on s’éloigne des grandes métropoles. Les chiffres sont édifiants : il y avait 20 % de diplômés de l’enseignement supérieur dans les territoires ruraux en 2020, contre près de 32 % en France France métropolitaine. Nous ne pouvons tolérer cette ségrégation territoriale qui mine notre pacte républicain. Cette inégalité territoriale frappe aussi la jeunesse rurale en matière d’accès à la mobilité. La Cour le rappelle, la première contrainte à la mobilité est non pas le prix, mais le manque d’offres de transport, notamment dans les zones périurbaines et rurales. Je citerai un exemple simple, mais parlant : 38 % des jeunes ruraux de 15 à 29 ans ont renoncé à un entretien d’embauche en raison de difficultés de déplacement. Construire une offre de déplacement pour la jeunesse dans les territoires moins denses meilleure coordination entre les autorités organisatrices de la mobilité, mais aussi des investissements. Les contraintes financières accrues pesant sur le budget des transports publics risquent de perpétuer les inégalités territoriales. Nos débats budgétaires sur le financement des mobilités seront donc cruciaux si nous voulons les résorber.

221 000 d’entre eux étaient accueillis et hébergés, dont plus de 31 900 jeunes majeurs. Là encore, les disparités sont frappantes. Certains départements mobilisent quatre fois plus de moyens que d’autres et le taux de prise en charge des jeunes issus de l’aide

46,3 % des jeunes âgés de 18 à 24 ans disaient avoir consommé au moins une fois dans leur vie du cannabis ; 3,5 % affirment en faire un usage quotidien

Oui, les pratiques récréatives à risque sont particulièrement répandues dans la jeunesse française. La Cour le rappelle : le repérage, l’accompagnement et la prise en charge des jeunes souffrant d’addictions font déjà intervenir la médecine de ville, l’hôpital et le secteur médico social, tandis que l’école

la figure de proue des publications de la Cour des comptes consacre cette année 612 pages au thème « Les politiques publiques en faveur des jeunes ». Monsieur le Premier président, vous avez déclaré que « la jeunesse représente les forces vives sur lesquelles repose notre avenir [et qu’] à ce titre elle est au cœur des préoccupations de nos concitoyens, ou du moins elle devrait l’être ». Tout est dans ces derniers mots : « ou du moins elle devrait l’être ». Ce rapport pose une question finalement simple : comment la France prend elle soin de sa jeunesse ? Le rapport chiffre à 53,4 milliards d’euros les dépenses de l’État en faveur des 15 25 ans. Ce budget, bien qu’il ne soit pas jugé excessif par la Cour, semble être mal ciblé et mal coordonné. Bourdieu disait que la jeunesse n’est qu’un mot. En effet, la jeunesse est une construction sociale, dans des univers sociaux qui n’ont parfois rien à voir. En ce sens, le rapport rappelle que les « jeunes » sont loin d’être une catégorie homogène. Il est salutaire que la Cour alerte sur leur exposition particulière aux inégalités de tous ordres – économique, géographique ou social. la jeunesse française expérimente peut être plus que d’autres que l’égalité des droits n’est pas celle des chances. À y regarder de plus près, on constate que plus d’un jeune de 15 à 25 ans sur dix est en situation de pauvreté, soit bien davantage que les 26 65 ans ou que les seniors. Le phénomène s’aggrave d’ailleurs depuis la fin des années 1960. Le rapport relève que les jeunes ont été « plus durement touchés que les autres catégories de la population par la crise économique provoquée par la pandémie » de covid 19.

Autrefois au cœur de la production du savoir et de l’enseignement supérieur, l’université publique française s’épuise désormais sous l’effet des injonctions contradictoires de la massification et de l’excellence. Les déterminismes y structurent encore trop souvent les parcours des étudiants et tant les grandes écoles que l’enseignement privé lui font concurrence. Pourtant, maintenir un haut niveau d’éducation

également le gel des recrutements des universités, qui anticipent de nouvelles coupes budgétaires, ou encore le limogeage de Katherine Calvin, la scientifique en chef de la Nasa.

la France doit pouvoir accueillir tous ces jeunes étudiants habitués à des conditions de recherche de haut niveau, qui contribueront au maintien de l’innovation française, dans un secteur très compétitif.

que le soutien public à l’accès au logement des jeunes non étudiants, majoritaires dans leur classe d’âge à compter de 21 ans, soit moindre. Les efforts menés par les pouvoirs publics depuis une dizaine d’années en faveur du logement jeune ont des effets limités.

Le constat d’une dégradation de la santé mentale des jeunes est apparu sur les radars du débat public pendant la pandémie. Depuis, rapports et missions d’experts convergent vers un diagnostic alarmant. Selon un baromètre publié en février dernier par Santé publique France, un jeune sur cinq présente des troubles dépressifs. S’y ajoute la hausse vertigineuse du nombre de passages aux urgences pour tentative de suicide, scarification ou empoisonnement volontaire, notamment chez les jeunes filles.

En effet, votre bilan des politiques publiques en faveur de la jeunesse n’est pas celui d’un échec complet. Il y a eu quelques réelles avancées, comme la hausse de 6 points du taux d’emploi des jeunes depuis 2017, le succès des politiques de mobilité ou encore la réduction de plus de treize mois des délais de jugement des mineurs.

La multiplicité des acteurs dont dépendent les financements et le choix d’une approche par sous populations cibles au détriment d’une approche globale rend impossible la mesure précise de l’investissement public ainsi que l’efficacité des actions menées.

Il en va de même du pass Culture, qui représentait 210 millions d’euros de dépenses pour l’État en 2023, sans aucun ciblage. Les inégalités sociales en matière d’accès à la culture demeurent.

avez vous identifié des perspectives de rationalisation des organismes et de clarification des compétences, notamment en matière d’orientation, d’accompagnement vers l’emploi ou encore d’aide au logement ?

Par lettres en date du 19 mars 2025, j’ai été informé par M. Dominique Théophile, vice président du Sénat, et par Mme Patricia Schillinger, secrétaire du Sénat, de leur souhait de démissionner de leurs fonctions respectives à compter du 31 mars 2025 à minuit. En conséquence, nous pourrions procéder à leur remplacement mardi 1 avril à